je vous remercie

Acte est donné de ces mises au point. Elles seront publiées au et figureront dans l'analyse politique des scrutins concernés.

Le montant de la prestation du cabinet de conseil McKinsey pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse s'élève à 957 674,20 euros. L'objectif est de préparer les transformations de la Caisse après la réforme des retraites. Sauf que ces prestations de conseil interviennent avant la réforme par points, abandonnée depuis De ces prestations, il ne reste rien ou quasiment rien : un et un carnet de cinquante pages qui ferait office de solde de tout compte. Monsieur le ministre, si des documents existent, il va falloir les communiquer largement à la représentation nationale, à la société civile et à nos concitoyens Sinon, il ne peut y avoir que défiance et suspicion. Je ne pourrai que vous le rappeler, en paraphrasant certains membres du Gouvernement plus prompts à enjoindre aux Français de travailler plus longtemps qu'à faire respecter les contrats des firmes privées : si tout travail mérite salaire, tout salaire mérite travail

Il a déclaré devant la commission des affaires sociales : « J'aurais été irresponsable si je n'avais pas pris le temps de me faire assister par une aide extérieure pour anticiper un tel choc. La Cnav a bien évidemment des compétences et des conseils en interne, mais pas pour absorber une telle transformation

que des conseils en stratégie. Je vous le demande, monsieur le ministre : des cabinets de conseil ont-ils directement ou indirectement participé à l'élaboration de la réforme des retraites dont nous discutons aujourd'hui ?

monsieur le ministre,

sans recours à des prestations de conseil. Les administrations, vous le savez, ont recours à ces prestations parfois sur des marchés structurants, parfois sur des marchés ponctuels, mais en l'occurrence, pour la préparation du PLFRSS que nous vous soumettons, le travail a été réalisé en interne. C'est d'ailleurs

dans ce qui existe déjà : je veux parler notamment des travaux du Conseil d'orientation des retraites (COR), lequel réunit toutes les grandes administrations concernées par ce sujet. J'ose le croire, si un jour était menée une véritable réforme des retraites, on commencerait par interroger ceux qui connaissent le sujet depuis longtemps !

en quoi avait consisté la prestation du cabinet de conseil McKinsey pour une somme de 957 674 euros, qui

M. Stéphane Le Rudulier. Depuis le début de l'examen de ce texte, on a souligné une réalité démographique implacable. Il faut rappeler les chiffres.

nous conduit à dire la vérité aux Français. Je crains fort que la mesure d'âge prévue à l'article 7, qui est nécessaire et indispensable pour préserver notre système de répartition, ne soit pas suffisante pour pérenniser définitivement le système auquel nous tenons tous ici, puisqu'il traduit la solidarité intergénérationnelle. C'est la raison pour laquelle, au travers de cet amendement d'appel, je demande au Gouvernement, avec bon nombre de mes collègues, de penser

évoquer une question de forme, monsieur le ministre. Il est bien dommage que vous ayez choisi une procédure rétrécie et très contrainte pour évoquer un dossier comme celui des retraites.

obligatoire de capitalisation, de provisionnement collectif- finalement une contribution de l'ensemble des salariés et des indépendants. Pourquoi ?

des systèmes de capitalisation. Vous venez de nous expliquer que c'est ce qui serait le plus juste pour les salariés. Pour notre part, nous disons que c'est ce qui serait le plus injuste et, surtout, le plus dangereux.

Qui pourra le faire ? Ceux qui le font déjà, c'est-à-dire ceux qui ont les revenus les plus importants. Demandez aujourd'hui à quelqu'un qui gagne le Smic ou même un petit peu plus d'économiser,

ce n'est pas un scoop, nous sommes contre la capitalisation, mais nous allons nous saisir de l'amendement de M. Husson pour essayer d'améliorer les choses et de vous montrer en quoi vous vous fourvoyez.

En 2019, les retraites s'élevaient à 288 euros en moyenne, avec une importante différence entre la pension moyenne des hommes et celle des femmes. Dans un pays où le niveau de vie est proche de celui du Portugal, les montants des retraites sont donc faibles et la plupart des personnes âgées doivent trouver un emploi informel pour subvenir à leurs besoins. système a été mis en place en 1981, sous la dictature de Pinochet, l'administration des fonds de pension était perçue comme un modèle novateur, qui faisait figure d'exception. Avant cette date, les Chiliens cotisaient à un fonds commun, géré par l'État, qui s'apparentait à un système de retraite par répartition. Aujourd'hui, ils déposent chaque mois environ 10 % de leurs rémunérations- salaires ou revenus imposables -sur un compte personnel auprès d'un administrateur de fonds de pension. L'objectif est que ces investissements produisent des rendements pour qu'à la fin de leur vie active les retraités puissent profiter à la fois du capital apporté et des gains accumulés. Malheureusement, le modèle chilien a montré ses limites. En 2018, l'OCDE considérait le Chili comme l'une des cinq économies mondiales au plus bas taux de remplacement. Autrement dit, un travailleur chilien qui part à la retraite subit une des plus grandes pertes de pouvoir d'achat. Pour ces raisons, nous demandons de mentionner cet exemple dans votre rapport : j'espère qu'il vous fera réfléchir.

d'un nouveau régime social applicable à des cotisations versées à un régime obligatoire d'assurance vieillesse par capitalisation destiné aux salariés et aux indépendants, régime qui serait intégré dans le système de retraite sans aucun débat démocratique avec les Français et les parlementaires, évidemment pas acceptable. Une telle modification du système de retraite ne peut se faire sans une consultation préalable du peuple. Définir une structure administrative qui pourrait être retenue pour piloter ce nouveau régime obligatoire, ses modalités de financement, la composition de son conseil d'administration, ainsi que les règles entourant les placements de ses actifs, donne évidemment l'impression que la réforme est déjà dans les cartons et dans les cartons et qu'il suffit d'une nouvelle majorité politique pour que cette réforme soit faite. Les auteurs de l'amendement justifient la pertinence d'une dose de capitalisation dans notre système de retraite l'exemple de l'Agirc-Arrco, alors que les cadres ont dû accepter une hausse de leurs cotisations salariales. Nous contestons l'introduction de la capitalisation dans notre système par répartition, dont les fondements reposent sur la solidarité entre les actifs et les retraités. Si la démographie modifie l'équilibre entre ces deux catégories, il faudrait augmenter la cotisation des employeurs pour garantir l'équilibre du système. Le sous-amendement

économiques (OFCE) : « Une génération qui remettrait en cause le système serait spoliée puisqu'elle devrait à la fois assurer une retraite à ses parents et se constituer un capital pour financer sa retraite par capitalisation. »

Ces deux amendements sont dans la droite ligne de ce que je soutiens depuis le début du débat : il faut introduire dans notre système de retraite une part réservée à la capitalisation.

Étudier ne devrait pas vous être interdit ! Comprendre le monde tel qu'il est ne devrait pas vous être interdit ! Voilà pourquoi j'ai déposé ces deux amendements

ils n'y sont jamais arrivés ! Aucun pays n'a réussi à tout unifier. Enfin, nous avons constaté que les systèmes de retraite de base étaient souvent des systèmes par répartition, mais que les systèmes complémentaires étaient gérés par les partenaires sociaux selon un système par capitalisation. Nous sommes les seuls en France

j'entends les défenseurs des sous-amendements affirmer qu'ils veulent limiter le champ du rapport à un certain nombre d'aspects pour ne pas ouvrir la question de la capitalisation,

tous, les premiers contempteurs des régimes par capitalisation sont souvent ceux qui par leur parcours personnel ont la possibilité d'avoir recours à un certain nombre d'assurances vie. Ces dernières, en fonction de la manière dont elles sont liquidées, ressemblent étrangement à des systèmes par capitalisation, dès lors qu'est fait le choix d'une rente mensuelle plutôt que d'un versement

mon explication de vote porte sur l'amendement n° 174 rectifié, puisque j'aurai ensuite une explication sur un autre amendement. Nous y voilà, chers collègues : il a fallu attendre le dimanche matin pour que le bâillon Retailleau se dénoue légèrement et que les masques tombent

Vous allez livrer la retraite des Françaises et des Français, fruit d'une vie de labeur, aux fonds de pension. Nous savons pourtant, vous et moi, que ces fonds sont des organismes sans aucune éthique. Ils se fichent complètement des enjeux environnementaux et sociaux dans le cadre de leurs investissements. Surtout, ils sont prêts à tout pour assurer le rendement de leurs placements. Vous allez donc siphonner les caisses du régime par répartition pour alimenter un système de retraite par capitalisation n'ayant pour effet que d'enrichir des investisseurs sans foi ni loi et de faire prendre des risques inconsidérés à notre régime de retraite sur lequel comptent nos compatriotes.

Vous faites donc le pari d'une société où la financiarisation continue à nous vider de notre substance et à vider le monde du travail de sa rémunération,

au travail par le capital. Voilà la réalité

en garde : à force d'insister sur la pénibilité de certains métiers, on finit par cesser de les rendre attractifs. Je vous suggère d'appliquer la recommandation de René-Paul Savary à la question des retraites ! À force de répéter aux jeunes que le système est plombé, on finit effectivement par leur faire perdre confiance. En fait, nous parlons moins des retraites

mauvais sens, mais celui des recettes. Vous avez élevé comme dogme depuis cinq ans le fait de ne pas augmenter les recettes et, au contraire, de les diminuer. Vous avez diminué le nombre de fonctionnaires, donc les recettes liées à leurs

a souligné à de nombreuses reprises les incertitudes liées aux marchés financiers. Il apparaît donc pour le moins paradoxal de vouloir sécuriser l'avenir de notre système actuel de retraite en le faisant évoluer vers un système mixte, intégrant un mécanisme qui soumettrait une partie de la retraite des Françaises et des Français aux aléas des fonds de pension et des fonds d'investissement. Par ailleurs, comme l'économiste Thomas Piketty, entre autres, a eu l'occasion de le souligner, le financement des retraites par capitalisation présente un autre risque, celui de l'aggravation des inégalités

Tout d'abord, le régime par répartition, qui était jusqu'à ce jour le meilleur, le plus généreux, est un régime redistributif-

de mondialisation libérale et de financiarisation. La capitalisation a permis de construire des acteurs financiers privés plus puissants que les États. BlackRock en est l'illustration la plus criante. Le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui la veuve du Michigan ou le boulanger de l'Ohio financent des projets qui les mettent eux-mêmes à genoux. Ils financent, d'abord, des projets climaticides,

ont altéré la rentabilité des placements financiers et provoqué une très lourde dépréciation des pensions. Comme le précise l'économiste Philippe Trainar, entre 1914 et 1939, les prix vont augmenter de 600 % au total, divisant par sept le pouvoir d'achat des rentes sur la période ». L'État français s'est alors tourné vers l'assurance publique et le système par répartition indexé sur les salaires

refuser d'aborder cette question de la capitalisation, c'est en priver les plus modestes ! La capitalisation

préfèrent partir nettement plus tôt, notamment ceux qui exercent des métiers difficiles- on revient à cette question de la pénibilité. Ils optent donc pour une formule qui leur octroie une pension réduite. Cette situation, conjuguée à une forte inflation-

je vous remercie

1 876 milliards d'euros de placements en assurance vie et 57 % d'entre eux sont propriétaires de leur logement. Croyez-vous que cette épargne ne soit pas destinée, avant tout, alors qu'il y a une certaine inquiétude sur l'avenir du régime par répartition, à consolider les moyens de nos compatriotes quand ils vont prendre de l'âge ? La capitalisation, ils la connaissent et la pratiquent, sauf lorsqu'ils n'ont pas les moyens d'épargner. Par conséquent, au moment où nos régimes par répartition- que nous nous efforçons de consolider sans beaucoup d'aide de votre part, chers collègues qui siégez sur la gauche

amener du provisionnement serait une manière de rétablir aussi la confiance dans la répartition. Ce provisionnement, nous en avons d'ailleurs la pratique. Le premier à l'avoir imaginé est M. Lionel Jospin : il n'a rien fait d'autre pour les retraites qu'un Fonds de réserve pour les retraites, comptabilisant aujourd'hui

en toute bonne foi à l'apport possible de la capitalisation pour renforcer la répartition

et de la majorité sénatoriale, qui le soutient. J'y vois la démonstration de votre volonté insidieuse d'utiliser la réforme initiale pour installer les conditions d'une migration progressive vers un système par capitalisation qui monterait en puissance dans les années à venir. Plus de sept Français sur dix rejettent votre réforme paramétrique fondée sur les 64 ans et les 43 annuités. Ils seront plus résolus encore et plus nombreux à rejeter la seconde réforme- cachée celle-là -introduite par ces demandes de rapport, y compris par le Gouvernement à l'article 1 , comme on le verra plus tard. Monsieur le ministre, pourquoi envisager la possibilité d'un système par capitalisation alors que vous nous présentez actuellement une réforme du régime par répartition ? Je constate que les composantes de la majorité sénatoriale sont toutes, sur le fond, favorables au système de retraite par capitalisation. Dans cette identité de vue avec la droite sénatoriale sur le fond, votre objectif cible, monsieur le ministre, est celui d'un système de retraite par capitalisation. Les Français doivent savoir que la réforme de la retraite à 64 ans n'est qu'une étape pour aller en ce sens. Plus la durée de cotisation au système actuel sera longue

J'ai entendu de l'autre côté de l'hémicycle dire que dans certains pays qui avaient choisi le système par capitalisation il était défiscalisé. Je tiens à préciser que le système par répartition repose sur des cotisations prises sur le salaire brut- cotisations patronales, cotisations salariales -et qui sont défiscalisées puisque la fiscalité s'opère sur le salaire net.

supplémentaires, paieront une complémentaire vieillesse sur leurs revenus. Voilà, c'est tout simple : on transpose à la vieillesse ce que l'on a déjà fait pour la santé.

Le moteur de l'étage suivant est alors allumé, la vitesse augmente. On place donc au sommet de la fusée ce que l'on veut emporter dans l'espace. Faire de la capitalisation le dernier étage de la fusée, c'est donc précisément faire de la répartition le premier étage à abandonner

Un modèle fondé sur la solidarité collective entre les membres de la société, dans le présent et entre les générations, et un modèle qui s'appuie sur la croyance absolue dans le fait que la spéculation financière, en soi, est une solution pour produire des richesses et pour mieux les répartir. Or qu'est-ce qu'a produit la spéculation financière ces vingt dernières années ? Elle a engendré les, la Grèce, la montée du prix des produits alimentaires de base. Au détriment de qui et au profit de qui ? Au détriment des plus pauvres et au profit de quelques grandes fortunes, qui- en plus ! -investissent dans des activités détruisant la solidarité, mais aussi la planète et, donc, notre capacité à avoir un monde dans lequel on pourra prendre demain une retraite

M. Le Rudulier a convoqué Jaurès dans cet hémicycle. J'aurais aimé que Jaurès s'exprimât lui-même, mais je vais lui prêter ma voix. Je le cite, dans C'est à l'invalidité que doit commencer la retraite. C'est au moment où ses forces diminuent que doit commencer la retraite du travailleur. » Tel est toujours notre projet. les retraites par capitalisation, vous avez dit quelque chose de très fort. Vous avez affirmé que le principal était la confiance : il faut avoir confiance dans un système de capitalisation.

vote. Je me pose une question depuis tout à l'heure, monsieur le ministre : le rôle d'un Président de la République est-il d'être le garant des fonds de pension ? Nous l'avons compris, vous avez une obsession qui ne vous quitte pas, vous et la droite sénatoriale : nous faire travailler plus longtemps, faire travailler nos enfants plus longtemps et les pousser à la capitalisation.

Maintenant on nous dit que ce régime ne peut être sauvé, sauf à capitaliser collectivement. Proposer un tel système, c'est affaiblir dans un premier temps la retraite par répartition- ça a été démontré - avant de le condamner complètement. Ce système par capitalisation reviendrait à nourrir des illusions dans la population, avec des promesses non tenues. Ma collègue a évoqué la situation des Chiliens. C'est, il est vrai, un exemple parfaitement éclairant. Difficile de parler de justice sociale et de capitalisation. Comment parler de solidarité générationnelle avec des placements, surtout au vu de leurs rendements ? Si la clé d'un régime par répartition est la démographie, comme j'ai pu l'entendre dire sur les travées de droite, celle de la capitalisation n'est en aucune façon la solidarité. solidarité. Au bout du compte, nous examinons un texte qui tend à fragiliser une grande partie de nos concitoyens. Comme si cela n'était pas suffisant, on veut leur enlever ce pourquoi on leur demande de contribuer toujours plus et encore plus longtemps ! La parole

: lorsque les Français investissent dans leur économie, ils garantissent la souveraineté du pays, notamment un bon déploiement de l'activité économique, au plus près de nos territoires.

financière. La répartition ne fonctionne- pour l'instant -qu'avec deux tiers des cotisations de retraite. Le dernier tiers, ce sont des impôts ou de la dette.

à notre système de retraite, on encourage les retraites parallèles avec des fonds de pension, ce qui remet en cause les fondements mêmes de la sécurité sociale. Le syndicaliste Régis Mezzasalma le souligne, ce système « pousse les salariés à réclamer des primes plutôt que des hausses de salaire, car ce sont les primes qui alimentent les plans d'épargne retraite ». Or, vous le savez, mes chers collègues, les primes sont exonérées de cotisations sociales. C'est une façon supplémentaire de siphonner notre sécurité sociale en épuisant les recettes de notre système. Cette politique libérale est le fil rouge de la politique voulue par le président Macron.

le Gouvernement proposait de travailler deux années complémentaires. Non, c'est la réforme Touraine qui allonge le délai à 43 ans. Quand vous commencez à 21 ans et que vous travaillez 43 ans, cela fait bien 64 ans.

permettez-moi de vous répéter qu'un système par répartition, par définition, doit être majoritairement composé de cotisations. C'est un système contributif.

Ce qui m'a amené à qualifier ainsi cette réforme, parfois à la surprise du président Kanner, dans un certain nombre de déclarations à la presse, c'est le fait que l'ensemble des gouvernements européens, qu'ils soient libéraux ou sociaux-démocrates, ont déjà procédé à ces réformes. La plupart des pays européens ont des âges de départ qui sont

Le scrutin est ouvert.

aussi que le pays, aujourd'hui, tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. » Et nous répondions à l'époque qu'effectivement « les distinctions sociales ne [pouvaient] être fondées que sur l'utilité commune ». Ces mots,

vous ne contribuerez pas à l'amélioration des retraites pour les plus modestes, en particulier les travailleurs dits essentiels.

86,9 jours par accident du travail, contre 79 jours pour les 40-49 ans. La durée moyenne d'un arrêt maladie est de 35 jours pour l'ensemble des salariés,

Le scrutin est clos.

à la même chorégraphie tous les sept ou huit ans, avec un certain nombre de réformes qui ont touché d'abord à la durée d'assurance, ensuite à l'âge légal. L'idée, c'est de commencer à préparer l'avenir,

Mme la rapporteure générale

la question des leviers. Certains prônent parfois des ajustements automatiques du système de retraite. Cette solution n'a pas ma préférence, dans la mesure où je pense que le Parlement, l'État et la classe politique doivent rester souverains en la matière.

sur l'article. L'article 1 fait référence à la réforme des retraites de 2019, laquelle visait la mise en place d'un système de comptes notionnels à cotisations définies et non plus à prestations définies. La différence est de taille : avec ledit système, le taux des cotisations sur salaire étant fixé une fois pour toutes, les droits à retraite peuvent être automatiquement et uniformément

sur les recommandations de Bruxelles. Dans ce système par points, les pensions sont la variable d'ajustement. S'il s'avère que l'espérance de vie moyenne augmente plus vite que prévu, si la conjoncture économique se dégrade et que les recettes diminuent, ou si les investissements financiers rapportent moins, alors les pensions diminuent. Les retraités ont vu leur pension diminuer trois fois- en 2010, 2011 et 2014 -, en application des règles de pilotage automatique prévues par la réforme.

attachés à notre système de répartition, qui garantit à toutes et à tous une pension de retraite dont le montant ne peut dépendre des aléas économiques. La parole

par répartition à prestations définies, au profit d'un calcul de points dont la valeur de service comme le prix d'achat ne sont définis qu'annuellement. Dès lors, le caractère redistributif n'est pas inscrit dans le mécanisme même de la retraite par points,

ne porte pas sur l'application d'une loi de financement de la sécurité sociale : il n'a donc pas sa place dans le PLFRSS, en application de l'article L.O. 111-3-12 du code de la sécurité sociale. Je crois que, sur ce point, nous serons tous d'accord

Il nous faut continuer à améliorer le système pour le rendre plus juste. En particulier, nous devons ensemble poursuivre la réflexion sur la convergence des régimes et des règles avec l'ambition de nous rapprocher d'un système de retraite plus universel.

Nous devons protéger le système de répartition pour la solidarité. Et je dénonce justement, monsieur le ministre, le fait que les cabinets de conseil vous alimentent en éléments de langage sans être efficients !

Pourquoi remettre ce sujet sur la table au détour du projet de loi dont nous discutons aujourd'hui si vous ne voulez pas présenter aux Français cette réforme voulue par Emmanuel Macron ?

mauvais rapports. Faisons le tri : celui-ci est extrêmement mauvais. L'article 1 dispose : « Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité, les conditions et le calendrier de mise en oeuvre d'un système universel de retraite faisant converger les différents régimes et intégrant les paramètres de la réforme prévue par la présente loi. » Tout est dit : ce dont nous débattons aujourd'hui n'est qu'une étape

aux conditions et au calendrier de mise en oeuvre d'un système universel de retraite. C'est la porte ouverte au régime de retraite par points, dit « universel », un projet que le Président de la République avait porté lors de son premier quinquennat. Les Français et les Françaises avaient massivement exprimé leur opposition à ce projet de réforme, mais vous avez de la suite dans les idées. Nous aussi, et les Français également ! Souvenez-vous de cette grève mémorable, à la fin de 2019 et au début de 2020, durant laquelle la SNCF et la RATP avaient battu le record des jours de grève

M. Delevoye, dont on n'a plus entendu parler depuis, M. Pietraszewski, dont j'avais moi-même oublié qu'il avait joué un rôle dans cette affaire ou encore Édouard Philippe, qui lui-même n'avait pas le même avis que le Président de la République sur ce sujet. Mais que sont-ils venus faire dans cette galère ?

qui n'a pas sa place dans un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. En l'espèce, le rapport prévu sur la mise en oeuvre du système universel de retraite n'a pas pour objet-

du système de retraite, fondée sur un régime universel par points. Cela entre en pleine contradiction avec le reste du projet de loi, qui met en oeuvre une réforme paramétrique portant sur l'âge d'admission à la retraite et le nombre d'annuités nécessaires. Le Gouvernement avait proposé un tel système en 2019, puis avait été contraint de le retirer. Le rapport proposé par l'intermédiaire de l'article 1 cherche à faire revenir par la fenêtre ce que nous avons fait sortir par la porte. Troisièmement, Troisièmement, cet article tend à rétablir l'unification du recouvrement social qui s'inscrivait dans le cadre du système universel de retraite.

le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur la possibilité, les conditions et le calendrier de mise en oeuvre d'un système universel de retraite faisant converger les différents régimes en intégrant les paramètres de la réforme prévus par la présente Veut-on suivre ici l'exemple suédois évoqué plus tôt dans nos débats et dont le résultat a été l'abandon du régime par répartition ? Le système suédois est aujourd'hui dénoncé par ceux-là mêmes qui l'ont mis en place.

Il me semblait, par ailleurs, que la Première ministre avait écarté la retraite par points voilà quelques semaines. Cet article n'a donc pas lieu d'être.

le recul de l'âge de la retraite et le glissement vers un système par capitalisation, soit une course à l'injustice sociale, au mépris des Françaises et des Français. Pour ces raisons, nous demandons la suppression de l'article

La suite, nous la connaissons. Nous l'avons tous lue dans le livre-enquête : c'est le scandale des méthodes de soins et de gestion du groupe Orpea, les maltraitances, les comportements négligents, la facturation de confort hôtelier hors de prix aux patients, mais aussi les pressions managériales

présentant le 10 janvier dernier une nouvelle réforme des retraites, cette fois-ci paramétrique, Élisabeth Borne semblait avoir signé elle-même l'arrêt de mort définitif de la retraite par points. Il n'y avait donc pas lieu d'agiter de nouveau le spectre d'une future mise en oeuvre d'un système universel de retraite intégrant, qui plus est, les paramètres de la réforme prévue par le présent projet de loi. Les Français ont clairement exprimé qu'ils ne voulaient aucune des deux réformes : ni celle de 2019 ni celle que vous nous présentez aujourd'hui,

pardon, mais il leur dit en plus que, pour le prix d'une réforme, ils en auront deux : le report de l'âge et le retour de la capitalisation. Les Français voient ces tergiversations de forme comme une provocation.

à finalité essentiellement budgétaire, déjà ! -d'un vernis systémique, en introduisant une discussion sur l'idée d'une retraite par points. Les Français ne s'y sont pas laissés tromper et ont massivement rejeté ce projet. L'état de l'opinion, puis l'urgence à l'épidémie de covid-19 ont ensuite contraint Emmanuel Macron à surseoir à ce projet. À l'évidence, si l'on en juge par ce nouvel article 1 , il n'y a pas renoncé.

un an après la promulgation de la loi, de la convergence des régimes de retraite vers un régime universel. Dans le dossier de presse portant sur le projet de loi actuel, il était indiqué : « Les régimes autonomes (professions libérales et avocats) et ceux répondant

Pourquoi le système par répartition a-t-il été préféré au système par capitalisation ? D'abord, parce que, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le système par répartition, fondé sur les cotisations, résout les questions de trésorerie et de réserves, particulièrement délicates au lendemain d'une guerre et d'une occupation qui ont ruiné le pays. Ensuite et surtout, parce que la capitalisation a montré ses risques et défauts. À l'époque, l'inflation va bon train. L'opinion ne croit plus aux rentes nominales, laminées par la hausse des prix. on veut dissocier le financement de la protection sociale de placements et de circuits financiers pour le moins incertains. C'est ainsi que le nouveau système s'impose.

les Français se prennent de passion pour notre travail. Ils nous écoutent et je ne veux donc pas passer mon tour ! Je souhaite donc également vous dire pourquoi cette proposition de rapport supplémentaire, sur une réforme qui viendrait modifier la réforme sur laquelle nous travaillons- c'est tout de même un paradoxe ! -, me semble inutile. Le régime de retraite par points, qualifié d'universel, a été rejeté massivement par les Français lors du

Le 10 janvier dernier, Mme la Première ministre a tiré un trait définitif sur l'idée d'une nouvelle réforme des retraites par points. Elle en propose une, que l'on qualifiera de

en oubliant la réalité de nos territoires et de la vie des Français, de nos concitoyens. Les partenaires sociaux et la grande majorité des Français refusent et refuseront encore cette opacité évidente.

Vous allez utiliser la réforme initiale pour installer les conditions d'une migration progressive vers un système par capitalisation. Après avoir rejeté le système dit universel en 2019, les Français s'opposent- vous le savez -à votre réforme paramétrique fondée sur un départ à 64 ans. Ils seront plus résolus encore à rejeter la seconde réforme, cachée celle-là, dont vous faites l'annonce, au débotté, par cet article. Pourquoi donc proposer ce rapport sur le système par points, alors que vous présentez actuellement une réforme des paramètres de notre régime par répartition ? Nous avons pu constater, ce matin, que les composantes de la majorité sénatoriale sont toutes, sur le fond, favorables au système des retraites par capitalisation. Dans cette identité de vue avec la droite sénatoriale, votre objectif cible, monsieur le ministre, est celui d'un système de retraite par capitalisation. Les Français doivent savoir que la réforme des 64 ans n'est qu'une étape pour aller dans ce sens. Plus la durée de cotisation au système actuel sera longue, plus le magot sera juteux pour les fonds de pension. Si cette voie est empruntée